et droits des services. Certaines communes sont très touchées par ces pertes de recettes tarifaires, notamment les petites communes rurales, qui ont plus souvent recours à des systèmes de régie pour la gestion de leurs services que les grandes villes.

une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement au titre de l'année 2020 mise en oeuvre sur délibération de la commune concernée. Cet amendement vise à intégrer les pertes ayant pour origine une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement au titre de l'année 2020

savons très bien quelles sont les méthodes de Bercy quand on veut compenser. Le meilleur moyen, pour Bercy, est de trouver un mode de calcul qui réduise au maximum la compensation. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas fait dans le passé

permettant à l'ensemble des AOM de bénéficier du dispositif prévu à l'article 5 du présent projet de loi, nonobstant l'hétérogénéité de l'organisation institutionnelle et financière de ces dernières. Ainsi amendé, ce dispositif constituera une première réponse aux difficultés financières rencontrées par les AOM doublement pénalisées par la baisse du versement mobilité et la chute de leurs recettes tarifaires. Il conviendra de traiter la question des recettes tarifaires dans un second temps, une fois établi le bilan économique précis, pour les AOM et leurs opérateurs, de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le financement des services publics de transport de voyageurs. Ce soutien aux AOM locales garantirait l'offre et la qualité de service des réseaux de transport, mais également les emplois directs et indirects de ce secteur

le produit moyen du versement mobilité entre 2017 et 2019, d'une part, et le produit de ce même versement perçu en 2020. Or cette disposition ne tient pas compte des spécificités des autorités organisatrices de la mobilité qui ont procédé, au cours de la période de référence, à une augmentation de taux et/ou à une extension de périmètre dans le cadre d'un projet structurant. Mme Van Heghe cite le cas du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle, qui vient d'achever un projet de transport en commun en site propre, avec une extension de périmètre, d'un montant de 400 millions d'euros, opération financée en grande partie par l'augmentation du taux du versement mobilité.

a connu une situation particulière du fait de la mise en place du Pass mobilité : il y a eu un phénomène de rattrapage

provoquent l'engorgement des marchés, la dépréciation de la valeur du bois, mais également l'absence d'exploitation et de débouchés du fait du ralentissement économique. La parole

La pandémie de covid-19 a généré divers problèmes, très préjudiciables à leurs recettes et ressources. La filière a été nettement bouleversée. Afin de soutenir ce service public de gestion des déchets qui est assurée par les collectivités territoriales, il est proposé ici, en raison

ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire, pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et des usagers. Pour celles qui financent ce service public une redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou une redevance spéciale pour les plus gros producteurs de déchets, il y a un risque important de perte de recettes en 2020. Il est donc proposé que les collectivités qui mettent en place le service public de gestion des déchets puissent également bénéficier de compensation pour ces pertes de recettes. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la redevance spéciale étant parfois instituées par les syndicats de gestion des déchets, il est également proposé que ce dispositif puisse leur être appliqué.

En effet, contrairement aux autres collectivités de France, la Guyane a connu en 2017 une crise sociale qui a eu un fort impact sur les recettes fiscales liées à la consommation et à l'activité économique en général. À titre d'exemple, les principales recettes fiscales de la collectivité territoriale de Guyane, la CTG, sont passées de 117,2 millions d'euros en 2016 à 108 millions Ainsi, on voit que l'impact de la crise est immédiat sur l'année en cours, mais il se poursuit encore sur l'année suivante, à savoir 2018. Ce n'est qu'en 2019 que le niveau de recette dépasse celui de 2016.

Enfin, la Guyane est une région qui connaît une très forte augmentation de population, avec des conséquences importantes en ce qui concerne les investissements en équipement : Saint-Laurent-du-Maroni, deuxième ville du territoire, doit par exemple créer seize classes d'école par an pour suivre l'accroissement de population. Cette croissance démographique rend également les recettes fiscales dynamiques, hors période de crise, ce qui signifie que, d'une année à l'autre, les recettes fiscales des collectivités connaissent normalement une croissance naturelle. plus la référence pour le calcul des pertes de recette est fondée sur des années éloignées, moins l'estimation des pertes sera juste et plus elle sera minorée, d'autant qu'elle ne tiendra pas compte de la croissance naturelle attendue.

à M. Georges Patient. Il s'agit d'individualiser chaque taxe pour la prise en compte de la variation de recette fiscale dans le calcul de la compensation à prévoir pour les communes d'outre-mer. Ainsi, ce sont les pertes réelles de chaque taxe qui seraient prises en compte, et non pas une moyenne des pertes, beaucoup moins proche de la réalité.

qui vise non pas sur la Guyane, mais sur l'ensemble des communes, départements et régions d'outre-mer, ses dispositions vont à l'encontre de la logique de compensation globale de l'article 5

La Guyane, c'est l'une des exceptions de la République : un territoire grand comme le Portugal, peuplé de 300 000 habitants, avec des difficultés immenses, car il a jusqu'à présent été considéré comme une simple position géostratégique de la France et une richesse pour l'Europe, avec le pas de tir de Kourou.

la moyenne 2017-2019 de l'octroi de mer communal en Guyane s'établit à 134 millions d'euros, tandis que les recettes d'octroi de mer de la seule année 2019 s'établissent à 113 millions d'euros. Et la DGG ! L'amendement n° 492 rectifié vise les seules communes. La moyenne 2017-2019 procède donc à un lissage avec l'année la plus faible, qui, pour les recettes communales d'octroi de mer en Guyane, est l'année 2019. C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré à M. Patient d'être attentif aux conséquences de cet amendement.

Le ralentissement de l'activité économique lié à la crise sanitaire a notamment entraîné une baisse importante de la consommation d'électricité, jusqu'à 20 % selon RTE. Cette baisse de la consommation aura un effet direct sur le produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, qui dépend de la quantité d'électricité consommée. L'article 5 du présent projet de loi vise à compenser pour les communes et les EPCI à fiscalité propre propre les pertes de recettes liées à la crise sanitaire, notamment pour cette taxe. Or cette dernière peut être perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre, mais également par les syndicats d'énergie et les départements, lorsqu'ils exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, ou AODE. Cet amendement vise donc à permettre également aux syndicats d'énergie et aux départements exerçant les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la distribution d'énergie de percevoir une compensation pour les pertes de recettes de TCCFE liées à la crise sanitaire. Le projet de loi prévoit déjà un dispositif permettant aux groupements de collectivités exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité de bénéficier des compensations pour les

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement considère que la consommation d'électricité des particuliers n'a pas spécialement évolué pendant la période de confinement et que seule la consommation d'électricité de grandes entreprises ou d'industriels a pu connaître de fortes baisses. Nous estimons donc qu'il est très peu probable que les syndicats d'électricité et les départements soient confrontés à une baisse importante de TCCFE en 2020. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas intégré cette taxe dans le dispositif de compensation. Par ailleurs, il faut avoir en tête que moins de cent syndicats exercent la compétence d'AODE et que plusieurs d'entre eux encaissent la taxe locale pour la reverser à leurs membres. Les inclure dans la compensation entraînerait un risque de double comptabilisation un travail de retraitement assez insécurisé techniquement et juridiquement, alors même que les syndicats ne subiraient pas de pertes en 2020. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable

chacun le sait, c'est 5 millions d'usagers des transports ; c'est la moitié du versement mobilité de toute la France ; c'est 60 % des utilisateurs du métro, du RER et des trains de banlieue.

C'est ce qui a conduit dans un premier temps, et encore aujourd'hui, le Gouvernement à proposer un traitement spécifique d'Île-de-France Mobilités, à ne pas le traiter comme les autres EPCI en charge de la fonction d'autorité organisatrice des mobilités.

en étant respectueuse des intérêts de chacun. J'ai même en tête, monsieur le rapporteur général, vos propos selon lesquels la vérité se situe certainement quelque part entre la position initiale du Gouvernement et la demande

C'est la raison pour laquelle, à ce stade, je le répète, le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Ce n'est pas une fin de non-recevoir ni une porte claquée, tant s'en faut. Il est juste absolument nécessaire de travailler de manière très approfondie sur un sujet qui, vous en conviendrez, est majeur budgétairement.

des amendements de la commission, mais attention : au-delà de la question de la compensation, cela signifie que, pour le moment, et en tout cas dans les mois qui viennent, la région ne pourra pas

Aujourd'hui qu'il est Premier ministre, je n'imagine pas un seul instant qu'il puisse revenir sur les engagements pris par le Gouvernement.

continuerons à utiliser des services dégradés faute d'investissements. Je n'imagine pas un seul instant comment Paris pourrait accueillir les jeux Olympiques dans ces conditions.

on sentait que les élections municipales étaient sous-jacentes dans les relations entre le Gouvernement et les parlementaires représentant ces territoires.

nous avons les plus grandes incertitudes sur la réalisation de ces équipements de transport lourds, pourtant nécessaires, notamment dans le cadre de la transition énergétique que nous appelons tous de nos voeux. Là

les parcs naturels régionaux sont des acteurs territoriaux reconnus. Concourant à la préservation de la biodiversité, ils sont gérés et aménagés par des syndicats mixtes. Le présent amendement vise à sécuriser l'éligibilité à la dotation prévue à l'article 5 pour les parcs naturels régionaux qui seraient touchés par des pertes de certaines recettes liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. Certes, les parcs naturels régionaux visés par l'amendement ont perdu des recettes tarifaires, mais ils n'ont pas perdu les contributions des membres. Je ne suis donc pas certain qu'il faille compenser l'ensemble des pertes de recettes, notamment parce que ces syndicats sont en France très largement financés

part, j'affirme que nous avons intérêt à afficher que l'ensemble du Sénat soutient la position du rapporteur général dans la CMP.

Elle est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires issues des dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, aux frais de formation des élus locaux élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Dans les petites communes, la moindre variation du potentiel fiscal peut avoir de lourdes incidences. Au regard de l'investissement considérable des élus des petites communes, notamment rurales, il est nécessaire que toutes les communes de 200 habitants et moins puissent bénéficier de la DPEL.

soient soldées à leur niveau de 2019. En raison de la prise en compte des recettes fiscales perçues en année-1 pour le calcul des contributions au FSRIF en année n, les collectivités qui contribuent à ce

85 est retiré.

Le droit à la consommation sur les tabacs représente pour les communes d'outre-mer la troisième rentrée fiscale fondée sur la consommation, après l'octroi de mer et la taxe spéciale sur les carburants. Les sommes en jeu représentent environ 260 millions d'euros pour l'ensemble des outre-mer. Il convient donc d'en tenir compte dans le calcul de la dotation visant à compenser les pertes fiscales des communes. D'après les premières estimations, fondées sur les quatre premiers mois de l'année, la baisse de recettes serait de l'ordre de 7 % à 8 %, soit environ 20 millions

compensation les recettes de l'octroi de mer et de la taxe spéciale de consommation pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, pour les collectivités uniques de Martinique et de Guyane, ainsi que pour le département de Mayotte. Le Gouvernement partage la position du rapporteur sur la question du tabac,

Malgré l'annonce d'une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal, le troisième projet de loi de finances rectificative tend à réduire artificiellement le montant des pertes en 2020. En effet, les pertes de recettes fiscales et patrimoniales sont calculées par comparaison non à l'année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Les montants obtenus sont ensuite réduits du montant des évolutions d'autres recettes fiscales locales. Enfin, le PLFR 3 ne comptabilise pas les baisses de recettes tarifaires, ni les dépenses engagées pour faire face à la crise. Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d'euros en 2020, alors que les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont à ce jour estimées, pour le bloc local, à 8 milliards d'euros sur trois ans, dont plus de 5 milliards d'euros En outre, le PLFR 3 abandonne le poids de la dette du covid-19 au contribuable local : son remboursement sera concentré sur les territoires les plus touchés par la crise sanitaire, et cette charge sera d'autant plus lourde que la collectivité a peu de marges de manoeuvre. Plusieurs voix ont d'ailleurs demandé la nationalisation des pertes de recettes et des dépenses engagées pour faire face à la crise. La virulence de la crise restant variable selon les territoires, la charge qui en résulte doit être supportée par la solidarité nationale pour éviter d'accroître les inégalités territoriales et permettre la participation des communes et de leurs EPCI au plan de relance. La parole est à M.

le rappelle, la DGG est calculée sur le produit global de l'octroi de mer, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement de la part versée

et à 109,5 millions d'euros en 2018. On remarque ainsi que l'impact de la crise est immédiat sur l'année en cours, mais qu'il se poursuit encore sur l'année suivante, à savoir 2018. Ce n'est qu'en 2019 que le niveau de recette dépasse celui de 2016.

M. Patient a raison sur les chiffres qu'il donne concernant l'octroi de mer pour la collectivité territoriale de Guyane. C'est ce qui a amené le Gouvernement, eu égard à la situation très particulière de la Guyane, à inscrire 8 millions d'euros de crédits pour neutraliser l'effet négatif que craint M. Patient si l'on ne prend en compte que la moyenne et pas de l'année 2019. L'inscription de 8 millions d'euros à l'Assemblée nationale pour neutraliser

Les recettes régionales éligibles à ce dispositif seraient les suivantes : la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ; la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ; l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ; l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre ; la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité

rencontrent aujourd'hui une situation difficile, compte tenu de l'absence de perception de la taxe de séjour au réel. Le présent projet de loi va renforcer le manque à gagner, puisqu'il prévoit la possibilité pour les collectivités de décider d'une exonération de la taxe de séjour, qu'elle soit au réel, au forfait ou mixte. De nombreuses collectivités ne pourront pas se le permettre. La cellule « tourisme » de la commission des affaires économiques estime qu'il convient, à titre tout à fait exceptionnel, de compenser la perte de recettes

Quel est l'avis du Gouvernement ? Le texte prévoit un mécanisme de garantie, qui inclut la taxe de séjour lorsque son produit baisse en raison de la diminution de fréquentation. Si une collectivité décide de diminuer la taxe de séjour, que ce soit en actionnant le droit commun

Cela étant, je souligne que le Gouvernement prend en charge une partie des dépenses liées aux équipements de protection individuelle. Je conviens bien volontiers que la discussion à l'Assemblée, puis au Sénat, a permis de compléter ce dispositif. Il faut aussi noter que le Gouvernement a inscrit, dès 2020, quelque 1 milliard d'euros de dotations supplémentaires pour accompagner l'investissement des collectivités. Enfin, j'ajoute que nous allons autoriser, par instruction comptable, la création d'un compte dédié pour les dépenses liées à la crise du covid, de manière à ouvrir aux collectivités un financement par

M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à élargir les dépenses éligibles au FCTVA aux dépenses d'équipements de protection individuelle,

S'agissant du taux, si le taux forfaitaire est actuellement de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1 janvier 2015, le présent amendement prévoit une augmentation du taux à 20 % sur les six prochains mois de l'année. S'agissant des dépenses éligibles, l'amendement vise un élargissement aux dépenses d'entretien des ouvrages d'art du périmètre des dépenses éligibles. S'agissant du remboursement, le présent amendement tend à généraliser le régime fondé

en effet à laisser aux collectivités territoriales leur capacité d'investissement. Il nous semble que le Gouvernement se doit de mobiliser de telles facilités budgétaires, surtout dans la mesure où il annonce un futur plan de relance. Un remboursement de la TVA sur les dépenses de l'année en cours irait dans ce sens, car cela

l'on réduit le délai de versement du FCTVA, les collectivités pourront accroître leurs dépenses d'investissement. La modification de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales permettra d'aller dans ce sens.

déjà présenté ici plusieurs amendements visant des évolutions liées aux finances locales à Mayotte. Ce territoire, vous le savez, a particulièrement souffert et continue à souffrir de la crise sanitaire.

Il représente la compensation forfaitaire versée aux collectivités et à leurs groupements pour la TVA qu'elles ont acquittée sur certaines dépenses d'investissement. d'investissement. Actuellement, le FCTVA est attribué au titre des dépenses d'investissements réalisées au cours de la pénultième année, n-2, de l'année précédente ou de l'année en cours. amendement vise à proposer une contemporanéisation du versement du FCTVA aux communes mahoraises, c'est-à-dire un versement des attributions du FCTVA l'année même de la liquidation de la dépense, comme pour les EPCI et pour les communes nouvelles de métropole. Cet alignement sur le régime, par exemple, des communes nouvelles aurait beaucoup de sens au regard de la structure des communes à Mayotte.

la question de l'anticipation ou de l'accélération du remboursement du FCTVA, l'amendement n° 1036 rectifié , auquel monsieur le rapporteur général apporte son soutien, est la redite du dispositif mis en place en 2009-2010 par Patrick Devedjian, qui était alors ministre de la relance.

c'est un fusil à un coup ! L'essentiel des collectivités, grâce à la disposition de 2009, est concerné par un remboursement à n+1. Si nous prévoyons un remboursement à n zéro, les collectivités auront un gain de trésorerie sur leur section d'investissement en 2020, mais nous ne pourrons plus procéder à la même opération ultérieurement.

rentrée. Je sais, en revanche, qu'en 2020 les sections d'investissement des collectivités dans leur ensemble sont globalement très bien financées, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'exercice 2019 s'est traduit par une amélioration de l'excédent de fonctionnement des collectivités, toutes strates confondues, ce qui se traduit par une augmentation du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement. Ensuite, 2020 est une année assez exceptionnelle pour le FCTVA, à hauteur de 7,6 milliards d'euros, ce qui est le fruit de la reprise de l'investissement en 2018 et 2019. Enfin, en 2020, nous disposons dans la loi de finances initiale

fait plutôt peser le risque d'une sous-consommation que d'une surconsommation des crédits. Dans la mesure où les sections d'investissement des collectivités sont bien équilibrées en 2020, et indépendamment du débat sur l'opportunité d'anticiper ou non en 2021 le remboursement de FCTVA, je considère que l'année 2020

la situation structurelle des communes de Mayotte. Vous le savez, après la départementalisation de 2011, il a fallu attendre 2014 pour que soit mise en place la fiscalité de droit commun. donc seulement à partir de cette date que les communes mahoraises ont commencé à être confrontées aux difficultés dont nous discutons aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai établi une comparaison avec les communes nouvelles.

sera sous-consommé s'il est utilisé pour faire de nouveaux investissements. S'il vient en abondement de la DETR et de la DSIL sur les projets en cours, il ne sera pas sous-consommé ; il viendra en support des finances et de la trésorerie des collectivités.

Par-dessus tout, la réforme de la fiscalité locale retire à ces collectivités le dernier levier fiscal sur lequel ils avaient un pouvoir de taux, en le remplaçant par une TVA sensible à la conjoncture. L'ironie du sort fait que nous le constatons aujourd'hui ... Le dispositif de compensation par des avances renouvelables est, certes, une bonne nouvelle, mais seulement à court terme, car les départements devront bien les rembourser, alors que leur avenir financier très incertain ; en outre, cela ne les encouragera pas ni investir ni à maintenir le niveau actuel des services publics. L'urgence nous appelle donc de vraies garanties aux départements, qui ne peuvent dépendre de prévisions hasardeuses quant à un éventuel rebond économique.

cette baisse de recettes en compensation. En revanche, le mécanisme, tel qu'il nous est proposé par le Gouvernement au travers de l'article 7- une avance sur droits de mutation remboursable relativement rapidement, même si l'Assemblée nationale a étalé ce délai

je trouve séduisante l'idée de la clause du retour à bonne fortune, je crains que l'adoption de cet amendement n'anticipe sur les discussions en cours avec l'ADF. Au cours de ces discussions, nous abordons bien évidemment

de 2014 à 2019, les DMTO ont augmenté de 5,5 milliards d'euros à l'échelon national, et le fonds de stabilité n'a été nourri qu'à hauteur de 120 millions d'euros, alors même que, en 2014, ce fonds avait été conçu

par rapport à leurs concurrents étrangers. Ainsi, cet amendement de notre collègue Jérôme Bignon vise à revenir sur ce déplafonnement, afin de conforter la compétitivité de nos industries. Quel est l'avis

Commençons par l'impact des amendements parlementaires adoptés en première partie. En premier lieu, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 1,5 milliard d'euros, compte tenu, notamment, de l'adoption de l'amendement qui tendait à élargir la liste des recettes éligibles au dispositif de dotation de compensation

En second lieu, les remboursements et dégrèvements d'impôts de l'État sont augmentés de 90 millions d'euros, ce qui dégrade d'autant le solde budgétaire. Cette hausse des remboursements et dégrèvements est liée, d'une part, à l'amendement qui visait à reporter au 1 janvier 2022 l'entrée en vigueur de la diminution du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et, d'autre part, à l'amendement ayant pour objet d'accorder un dégrèvement exceptionnel de contribution à l'audiovisuel public aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie.

notamment sur des mesures de relance, en particulier en faveur des entreprises. Je ne vais pas les détailler, car vous les connaissez tous. Je pense au report en arrière des déficits, dit « », à des amortissements accélérés,

chiffrent en milliards d'euros. Peut-être pour des raisons politiques, vous n'avez pas souhaité, à ce stade, compte tenu du tempo qu'a choisi le Gouvernement, afficher que le Sénat avait agi pour la relance. Vous vous êtes borné à

je rappelle que, en application de l'article 42 de la loi organique du 1 août 2001 relative aux lois de finances et de l'article 47 , alinéa 2, du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances rectificative, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous apprêtons à examiner les missions budgétaires, qui regroupent notamment les crédits que le Gouvernement souhaite mobiliser en soutien à l'industrie automobile.

Une grande partie de l'emploi industriel français en dépend. Le plan de soutien doit permettre aux entreprises de passer le cap de cette double crise d'offre et de demande, pour qu'elles puissent continuer à se concentrer sur les défis du futur : mobilités alternatives, véhicules autonomes, nouvelles énergies et, si j'ai bien compris ce qui a été dit ce matin, véhicules beaucoup moins lourds. C'est parce que ces défis sont immenses et incontournables que les aides que nous autorisons doivent avoir un caractère fortement incitatif. Ne versons pas de l'eau dans le sable et gardons à l'esprit un mot d'ordre : l'efficacité de l'action publique et des dépenses publiques. Monsieur le ministre, quelles contreparties avez-vous obtenues de la filière automobile avant de lancer ce plan de soutien de grande ampleur ? Nos dépenses publiques serviront-elles bien au maintien sur notre territoire de la production et des emplois ? Les entreprises relocaliseront-elles ce qui peut et surtout ce qui doit l'être ? Comment assurer que le renforcement du capital et les prêts de trésorerie auront pour finalité l'investissement dans l'avenir, et non la rémunération des actionnaires- y compris l'État -, parfois gourmands, ou le transfert vers des sites étrangers ? La recherche et développement et l'innovation s'orienteront-elles vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les énergies plus propres, sans se limiter à l'électrique ? Quel bénéfice notre industrie française tirera-t-elle des millions engagés dans l'Alliance européenne pour les batteries ? Je m'inquiète un peu du manque de transparence sur ces sujets. Le « quoi qu'il en coûte » ne peut s'entendre que s'il sert nos intérêts collectifs et comporte les garanties appropriées. Les engagements pris, par exemple, par Renault seront-ils rendus publics ? Comment surveillerez-vous leur respect

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous en arrivons à l'article 9 et à l'examen des ouvertures de crédits dans le budget général de l'État. Avant que nous examinions les quelque 170 amendements déposés sur cet article, je veux m'arrêter un instant sur l'hétérogénéité de ce troisième PLFR. mêlent saupoudrage budgétaire et planification catégorielle, au bénéfice de quelques secteurs et à l'exclusion de tous les autres. Nous y reviendrons lorsque nous étudierons l'article 18. Là où les deux premiers PLFR limitaient limitaient les ouvertures de crédits à quelques politiques publiques essentielles, ce troisième budget rectificatif ouvre des crédits dans pas moins de dix-sept missions du budget de l'État. On fait comme si la nécessité de la dépense publique était établie, sans tenir compte des capacités du pays à la financer. Je m'inquiète du déficit colossal que nous atteignons- près de 225 milliards d'euros -et du fardeau que nous allons transmettre aux générations futures, futures, ce d'autant plus que, sur les 40 milliards d'euros des plans sectoriels annoncés dans le PLFR 3, plus de 36 milliards d'euros sont reportés sur les années 2021 et suivantes. L'incidence de ces plans sur nos comptes publics sera donc massive dans les années à venir. L'emballement des dépenses publiques ne fait que commencer. La multiplication des plans sectoriels me paraît dangereuse. Elle est nécessairement arbitraire : la situation des entreprises est en réalité très disparate au sein d'un même secteur. Surtout, elle nourrit l'illusion de l'argent gratuit et encourage chaque secteur à se manifester à son tour pour réclamer tous azimuts sa part du butin, son propre plan Marshall. Cette approche ne peut que susciter la désillusion de ceux dont les revendications ne pourront être satisfaites.

Pris par le haut, tous les sujets deviennent des objets de posture ou de division. Sur le papier, on n'en fait jamais assez ! » Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion sur le périmètre du champ d'intervention de l'État. De grâce, définissez vos priorités ! Je suis saisi

L'article 9 prévoit l'ouverture de 1 milliard d'euros de soutien à l'investissement au titre des exercices 2020 et 2021, afin d'accompagner l'émergence de projets de territoires structurant localement et favorisant la coopération entre les acteurs locaux et étatiques. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti. Toutefois, fléchée sur des priorités fixées depuis Paris, elle ne permettra pas de répondre à l'ensemble des besoins. des territoires ruraux (DETR) soit également abondée, la priorité devant être donnée au soutien aux petits commerces de proximité, actuellement en grande difficulté. Nos territoires ruraux ne doivent pas être oubliés. Les projets d'accessibilité aux soins, la redynamisation des le développement de l'attractivité des communes de nos terroirs doivent aussi faire partie de nos priorités en termes de soutien à l'investissement. Il est ainsi proposé d'inclure proportionnellement aux crédits initiaux cette nouvelle dotation de 1 milliard d'euros au sein des enveloppes consacrées à la

Certains disent que c'est cher, très cher. Ils laissent sous-entendre que certaines gabegies expliqueraient les difficultés actuelles de ce réseau. Sans doute des injustices doivent être corrigées, mais le problème majeur de l'enseignement français, c'est d'abord un sous-financement de l'État,

Ils sont largement plus élevés qu'à l'étranger. Mais, à l'étranger, ce sont les familles qui les paient ! Et avec leur augmentation, le poids des frais de scolarité est de plus en plus significatif. Afin de maintenir une cohérence à ce réseau, il est essentiel de doter correctement l'opérateur qu'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour accompagner les établissements. C'est la manière la plus efficace de répondre aux besoins, et c'est encore plus indispensable en période de crise. La situation actuelle, nous la connaissons : des établissements sont fermés parfois depuis le début du

Dans ces conditions, il est très probable que de très nombreux établissements devront faire face à de grosses difficultés financières et perdront énormément d'élèves. Le plan qui a été prévu,

est l'avis du Gouvernement ? Gérald Darmanin et moi-même avons discuté avec Jean-Yves Le Drian d'un plan qui se traduit par des ouvertures de crédits dans ce PLFR. Nous savons que, sur certaines lignes- je ne dis pas toutes -, il y a quelques économies de constatation. Nous savons aussi que, en fin de gestion, si c'était nécessaire,

des frais de scolarité. Or qu'en était-il quand François Hollande est arrivé au pouvoir ? J'ai le rapport de Claudine Lepage : à l'en croire, le

Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de crédits supplémentaires. En effet, une enveloppe de 50 millions d'euros d'aide exceptionnelle a déjà été votée pour venir en aide aux Français en difficulté.

L'objet de cet amendement est d'autoriser qu'une partie de l'enveloppe de 50 millions d'euros- à savoir 10 millions -soit fléchée sur les Français qui ont créé leur propre petite entreprise, en leur accordant, sur dossier évidemment, six mois de trésorerie pour leur permettre de redémarrer.

des entrepreneurs français à l'étranger. C'est un point que nos services doivent suivre, y compris au titre de l'aide sociale, au vu de l'hétérogénéité de la situation des entrepreneurs et de la difficulté que nous aurions à mettre en place une intervention de nature économique, les comptabilités et les références auxquelles ils sont soumis étant, par nature, très différentes.

que toutes les conditions que Bercy a imposées pour ouvrir droit à ces crédits soient levées et que ces 50 millions d'euros puissent effectivement être utilisés le mieux possible par les conseillers des Français de l'étranger,